La rédaction actuelle place hors du champ de cette exonération les ventes aux aménageurs publics ou privés, lesquels ne créent pas les logements sociaux alors qu'ils ont vocation à préparer les fonciers destinés à les accueillir. le même particulier qui vend un terrain à un aménageur, lequel viabilise un terrain en vue de la réalisation de logements sociaux, cesse d'être éligible à cette exonération d'impôt. Cela affecte la concurrence au préjudice des aménageurs publics et privés. est donc proposé : d'une part, d'étendre le champ de l'exonération de plus-values immobilières aux cas de cession par un propriétaire particulier en fonction de la destination du bien immobilier, c'est-à-dire la production de logements sociaux, indépendamment du statut de l'acquéreur ; d'autre part, de fonder le calcul de l'exonération, à partir de la surface

qui précise les modalités d'application de l'exonération sur les plus-values immobilières lors d'une cession à un organisme de logement social. L'amendement ne peut donc être accepté. J'en demande le retrait.

il n'y a pas véritablement de raison de faire de différence et de priver le vendeur de l'exonération sur les plus-values, à partir du moment où on est certain qu'au bout du compte on construira du logement social. Néanmoins,

À partir du moment où le propriétaire vend et qu'il y aura construction de logements sociaux, que ce soit un aménageur qui achète en premier ou directement un bailleur social, quelle que soit sa forme,

très restrictive par rapport au dispositif qui existait auparavant. Elle conduit, en effet, à supprimer l'application de ce régime dans le cas où l'organisme destine le bien acquis à une opération d'accession sociale à la propriété ou encore à une opération telle que la construction de centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Par le présent amendement, nous proposons donc d'élargir l'affectation aux principales opérations de logement social constituant le service d'intérêt économique général confié aux organismes de logements

Pour encourager la création de logements sociaux, l'article 150 U du code général des impôts accorde une exonération d'impôt sur les plus-values au bénéfice des personnes physiques lors des cessions d'immeubles au profit soit d'organismes de logements sociaux, soit d'opérateurs qui s'engagent à réaliser des logements sociaux. L'intention du Gouvernement est de recentrer le dispositif sur le logement social, mais l'interprétation retenue est extrêmement stricte. Elle conduit à supprimer l'application de ce régime aux cessions de terrains destinés à une opération de logement en location-accession et à une opération logements en bail réel solidaire (BRS). Nous proposons de réintroduire ces deux catégories de logements assimilés à des logements locatifs sociaux par l'article 55 de la loi du par ailleurs, d'élargir la liste des organismes éligibles pour inclure les organismes de foncier solidaire qui portent les opérations de bail réel solidaire. Le dispositif BRS est devenu l'outil anti-spéculatif des collectivités qui veulent agir au service de l'accession à la propriété des ménages à revenus modestes. Il a vocation à se développer sur tous les territoires, dès lors qu'il y a un enjeu de maîtrise du foncier. Certes, il existe la possibilité d'un abattement de 75 % s'appliquant aux produits de cession, mais il fonctionne uniquement dans les zones tendues. Or les opérations réalisées dans le cadre d'un bail réel solidaire ne sont pas toujours en zones tendues et doivent pouvoir se mettre en place partout sur le territoire. Cette proposition est en cohérence avec les programmes de soutien aux petites et moyennes villes, comme « Action coeur de ville et « Petites villes de demain ». Le bail réel solidaire est l'une des solutions qu'il faut absolument développer pour permettre le logement abordable. Nous proposons donc de soutenir les organismes de foncier solidaire qui ont besoin de foncier pour déployer leur activité sur l'ensemble du territoire. Plus globalement, tout ce qui vise à favoriser la construction de logements sociaux neufs doit être mis

bénéficient d'une exonération d'impôt pour les plus-values. L'article 3 en précise les modalités, en indiquant notamment que l'exonération ne s'applique que dans la mesure où l'organisme s'engage à réaliser des logements sociaux

intervient dans un montage où un ménage modeste peut accéder à la propriété de manière progressive ; l'OFS demeure propriétaire du terrain, ce qui permet de réduire le coût de l'acquisition pour le ménage, en garantissant que le prix de cession restera modéré sur le long terme, lorsque le ménage le revendra. Les opérations d'accession sociale à la propriété bénéficient, d'ailleurs, de certaines exonérations fiscales et d'aides de l'État, par exemple le taux réduit de TVA à 5,5

proposent d'étendre cette liste à la plupart des opérations relevant du service économique d'intérêt général du logement social. Les auteurs des amendements identiques n I-36 étendent la liste aux logements en accession à la propriété ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire. La deuxième série est plus précise. J'émets donc un avis favorable sur les amendements identiques n I-36 rectifié

permet de rapprocher les régimes applicables aux opérateurs privés et aux organismes HLM et assimilés en matière de cessions d'immeubles. Nous soulignons qu'elle n'empêche pas l'exonération totale de la plus-value lorsque les organismes HLM réalisent des opérations autres que la production de logements destinés à la location sociale, mais qu'elle restreint simplement leur part à 20 % des programmes. Nous ne sommes donc pas favorables aux extensions de l'exonération aux seuls organismes de foncier solidaire pour leur permettre de réaliser des opérations de location-accession à la propriété. Nous ne sommes pas non plus favorables aux autres dispositions proposées par les amendements. Le Gouvernement est donc défavorable à la totalité de la série

celui qui vend. Car l'avantage doit être pour le propriétaire qui, au moment de céder son terrain, doit être incité à faire le choix d'un cessionnaire qui construira du logement social.

lors des cessions d'immeubles au profit d'organismes de logements sociaux ou d'autres cessionnaires qui s'engagent à réaliser des logements sociaux. Il ne concerne néanmoins que les constructions neuves

? L'exonération a pour objet de favoriser les logements sociaux. Il est donc normal que, dans le cas d'un programme mixte, elle s'applique au prorata de la surface consacrée aux logements sociaux : c'est l'un des principaux apports de cet article par rapport au droit existant. Le débat porte ici sur la manière dont est calculée la surface des constructions l'article 3 indique que c'est la surface mentionnée sur le permis de construire, ce que cet amendement conteste au motif que le permis de construire est susceptible d'être donné plusieurs années après la cession- En effet l'organisme de logement social dispose de dix ans pour construire les logements, mais l'exonération s'applique dès la cession. Cet argument paraît fort, mais j'observe que, dans le droit existant, la surface prise en compte est déjà celle du permis de construire dans le cas où c'est un cessionnaire autre qu'un organisme de logement social qui s'engage à construire les logements sociaux. Dans ce cas, cet amendement reviendrait sur le droit existant. Je Je propose donc de recueillir l'avis du Gouvernement pour voir s'il faut améliorer ce point de rédaction de l'article 3 : peut-être faudrait-il, par exemple, que la surface de logements sociaux réalisés soit mentionnée sur l'acte authentique d'acquisition et non sur le permis de construire.

que le cessionnaire s'est engagé à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnée sur le permis de construire. Supprimer la référence au permis de construire priverait la réforme d'efficacité, dès lors qu'il ne serait plus possible d'apprécier le pourcentage de logements sociaux au regard de ce critère objectif. Je retire l'amendement, monsieur le

parole est à M. Thierry Cozic. Afin de répondre aux besoins exprimés dans le cadre du plan Logement outre-mer et compte tenu du contexte de crise, le présent amendement vise à prolonger de deux ans le dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer en faveur des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements libres, qui doit s'éteindre au 31 décembre 2020. En outre, cet amendement vise à assouplir la condition d'ancienneté du logement pour bénéficier du dispositif, en la portant à quinze ans, afin de tenir compte du vieillissement accéléré des logements outre-mer

à ces amendements, puisque le dispositif est d'ores et déjà prolongé par un article adopté en seconde partie du présent PLF.

Je rappelle que les dispositifs de défiscalisation outre-mer en matière de logement répondent à des difficultés spécifiques : habitat insalubre, nombre insuffisant de logements, notamment sociaux. Des travaux Des travaux d'amélioration ou de rénovation ne répondant pas directement à ces objectifs de politiques publiques me semblent trop larges. Enfin, des dispositifs prévoient d'ores et déjà des mécanismes particuliers pour la réhabilitation ou la confortation contre le risque sismique et cyclonique.

pour les investissements réalisés outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d'agrément préalable, ce statut d'associés limitant l'engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société.

à ses associés commanditaires pour les investissements réalisés outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d'agrément préalable, ce statut d'associés limitant l'engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société.

tend en réalité à étoffer la nature des dépenses éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt en faveur des investissements dans les logements situés en outre-mer et affectés à la résidence principale. Je précise que le Gouvernement est favorable à la prorogation de la réduction d'impôt en faveur des travaux de réhabilitation et de confortation contre les risques sismiques et cycloniques, telle qu'adoptée à l'article 42 C du présent projet de loi. Or l'adoption de l'amendement aurait pour effet de modifier en profondeur le champ de réduction d'impôt outre-mer, en l'étendant à des dépenses déductibles des revenus fonciers,

au service de location de vélos et de trottinettes à assistance électrique ou de scooters électriques en libre-service, qui aura du mal à se développer en outre-mer sans l'appui de l'aide fiscale, compte tenu des handicaps structurels de ces territoires.

outre-mer, où le maillage du réseau de transports collectifs est encore largement insuffisant et le réseau routier quotidiennement saturé, le besoin de solutions nouvelles pour une mobilité durable est devenu primordial. Le présent amendement vise donc à ouvrir la liste des secteurs bénéficiant du champ de l'aide fiscale à l'investissement qui en sont aujourd'hui exclues, et plus précisément au service de location de vélos et de trottinettes à assistance électrique ou de scooters électriques en libre-service, qui aura du mal à se développer en outre-mer sans l'appui de l'aide fiscale, compte tenu des handicaps structurels de ces territoires.

particulièrement exposé à la concurrence internationale. Pour l'essentiel, le secteur tertiaire en est exclu, raison pour laquelle l'avis est défavorable.

Les besoins demeurent très importants, y compris en matière de rénovation et de réhabilitation hôtelière. La crise sanitaire vient doublement éprouver le secteur hôtelier. Il convient donc de renforcer l'attractivité des investissements par la fiscalité, en portant le taux de réduction d'impôt, actuellement établi à 45,9 %, à 53,55 %.

son territoire du taux de droit commun. Il est inexplicable, alors même que les difficultés sont indéniables, que le taux de réduction soit inférieur au taux de droit commun. Nous ne comprenons pas l'entêtement du Gouvernement.

prévue aux opérations de reconstruction de logements et à supprimer la condition d'ancienneté du logement pour son bénéfice, à la condition que les territoires et communes

est défavorable, car le mécanisme de réduction d'impôt prévoit déjà un ensemble d'outils qui permet le développement et la rénovation du parc locatif social dans les collectivités d'outre-mer. Nous insistons sur le fait que les mécanismes de défiscalisation outre-mer en faveur du logement répondent à une logique de programmation selon les besoins des différentes collectivités, pour satisfaire des besoins structurels, et non conjoncturels. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement de Saint-Martin, l'État a tenu ses engagements dans le cadre de la reconstruction de cette collectivité. Je pense notamment aux fonds mis à disposition, même si, évidemment, le travail reste important sur place. Quel est donc l'avis de la commission ?

notamment en raison de la petite taille des systèmes électriques des ZNI, qui ne permettent pas d'opérer des économies d'échelle afin de rendre les marchés locaux plus rentables. Afin d'équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l'ensemble du territoire national les charges financières liées à la contribution au service public de l'électricité pesant sur le consommateur. Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d'égalité devant l'impôt. Le Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n'interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI pluriannuelles de l'énergie (PPE) spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique. Leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié. Quel est l'avis de la commission

production d'électricité qu'elles connaissent, cette solidarité représentera plus de 2,6 milliards d'euros sur le budget de l'État en 2021. Il ne me paraît donc pas souhaitable de prévoir des aides supplémentaires

les travaux de reconstruction sont toujours en cours. Si le fonds d'urgence pour le logement, supprimé par la loi de finances pour 2020, a contribué à la prise en charge des sinistrés de l'ouragan sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, et a notamment apporté une dotation exceptionnelle de 6 millions d'euros à la collectivité de Saint-Martin, force est de constater que la partie française de Saint-Martin

du crédit d'impôt en faveur du logement social en outre-mer. Cependant, celui-ci ne constitue pas le vecteur adapté pour Saint-Martin, dans la mesure où ce territoire bénéficie d'une autonomie fiscale et d'une fiscalité locale propre. De manière générale, une société une société ne peut se voir appliquer un crédit d'impôt sur un territoire à compétence fiscale propre : il faut payer des impôts sur le territoire français dans le régime de droit commun pour en bénéficier. C'est une constante de notre droit fiscal.

Or il existe aujourd'hui une tension très forte sur la programmation des PLS pour 2021, qui devrait perdurer dans le temps. Il est fort probable que certaines opérations soient reportées. D'autres devraient évoluer vers du locatif intermédiaire pour les investisseurs institutionnels. Dans ces conditions, le présent amendement tend à rehausser de 10 points le quota actuel de logements PLS dans les départements d'outre-mer.

de favoriser la construction de logements sociaux et très sociaux outre-mer. Il est normal que le logement intermédiaire, dont font partie les PLS,

Cependant, les ménages qui y habitent ont des capacités contributives limitées et une faible capacité à pouvoir accepter une augmentation des loyers après leur réhabilitation. Il s'agit de favoriser les réhabilitations hors quartiers politique de la ville à moindre coût.

NPNRU, 34 se trouvent dans les départements et régions d'outre-mer : 5 en Guadeloupe, 3 en Martinique, 14 en Guyane, 4 à Mayotte et 8 à La Réunion.

Aujourd'hui, le code général des impôts permet aux organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer de bénéficier d'un crédit d'impôt. Celui-ci est notamment valable pour les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs, lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. De plus, lorsque l'investissement revêt

de prolonger le délai des chantiers si l'opération dépasse deux ans, selon des conditions et modalités définies par décret.

rectifié, il me paraît normal que les délais de construction soient encadrés, ce qui permet d'ailleurs de protéger les investisseurs contre des opérations trop longues.

logement social. Le bénéfice du crédit d'impôt s'applique à une opération de construction ou de réhabilitation sur un logement social. Ces opérations consistent en des investissements et en une déclinaison opérationnelle longue, qui peut atteindre quarante le bénéfice est comptabilisé sur la seule première année, faussant ainsi les comptes de l'organisme de logement social (OLS), qui affiche un résultat exceptionnel, tandis que son résultat sera largement négatif sur toutes les années suivantes du déploiement de l'opération. Cette hypothèse peut conduire à un défaut de validation des comptes des OLS par les commissaires aux comptes, ce qui les empêchera d'assumer leur activité. Afin de permettre une lecture juste des comptes des organismes de logements sociaux, il est nécessaire que le bénéfice du crédit d'impôt s'étale, comptablement, sur toute la durée de l'opération, ainsi que c'était le cas avec la défiscalisation.

ce dernier dispositif peut précisément faciliter la reprise ou la restructuration de l'entreprise concernée, certains investissements étant susceptibles d'entrer dans le plan de réorientation ou de rationalisation de son activité.

-dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d'une procédure de mandat de conciliation de conciliation ou de sauvegarde de l'entreprise exploitante. Dans la mesure où les aides aux entreprises en difficulté ne sont pas couvertes par le règlement général d'exemption par catégorie, la conformité au droit européen de l'extension proposée du champ d'application de l'aide fiscale nécessite une autorisation individuelle systématique de la Commission européenne.

de précaution (DEP), nouveau levier fiscal plus efficient réservé aux entreprises imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d'imposition. Les entreprises agricoles relevant du régime d'imposition sur les sociétés en sont donc exclues, alors qu'elles sont sujettes, dans les mêmes conditions, aux aléas climatiques ou économiques et à la nécessité de constituer des réserves de précaution.

reste réservé aux entreprises imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d'imposition, ce qui exclut de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d'imposition sur les sociétés.

entre les différentes sociétés soumises à ce même impôt. Par ailleurs, cette mesure ne nous paraît pas justifiée, les entreprises agricoles soumises à l'IS étant imposées à un taux proportionnel et bénéficiant de la trajectoire de baisse de cet

d'immeuble. La prolongation du délai de quatre ans prévu par l'Assemblée nationale pour réaliser les travaux de transformation en logement des biens acquis est une bonne chose en temps de crise. Elle peut être justifiée par la complexité du chantier ou par toute autre situation exceptionnelle, en particulier dans le contexte sanitaire actuel. Une prorogation annuelle renouvelable de façon illimitée risquerait d'ouvrir des délais de construction très supérieurs aux quatre ans initialement prévus, ce qui nuirait à l'objet même de ce dispositif, à savoir la construction rapide de logements dans les zones qui en ont le plus besoin. Pour ces raisons, nous proposons de maintenir la prolongation du délai d'un an

Pour la même année, le délai médian atteint 22,7 mois contre 22 mois en 2018 et 19 mois en 2017. Cet amendement vise donc à encourager l'accession sociale en incitant les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logements à mieux répondre à la forte demande d'attribution de logements sociaux, en particulier dans les zones tendues.

l'avis du Gouvernement ? Le secteur du logement social profite donc de dispositifs d'incitation. Les cessions ayant pour objet la transformation en logements, notamment sociaux, d'immeubles commerciaux bénéficient d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés. La prorogation de ce dispositif n'est pas

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article, introduit à l'Assemblée nationale, tend à relever le montant du chiffre d'affaires en deçà duquel les petites et moyennes entreprises bénéficient du taux réduit de l'impôt sur les sociétés.

Vous le savez, nous défendons la justice fiscale pour les ménages. Nous considérons que les plus aisés doivent davantage contribuer à l'économie réelle. Notre logique est la même pour les entreprises nous souhaitons que la charge fiscale soit justement répartie. Les grandes entreprises, les multinationales qui disposent de moyens économiques conséquents doivent être davantage mises à contribution. Les PME et les TPE doivent bénéficier d'une baisse de l'imposition. Les PME de nos territoires et les commerces de proximité ont été fortement impactés par la crise sanitaire. Nos TPE et PME ont subi le confinement, le couvre-feu et maintenant un second confinement. un second confinement. Les PME doivent pouvoir évoluer dans un environnement favorable. Nous voulons leur redonner confiance. Les élus de la Nation doivent entendre les difficultés de nos PME. Soutenir ces dernières, c'est soutenir notre tissu économique. Elles doivent être défendues, et elles le seront par les sénateurs socialistes. Nos collègues de la majorité sénatoriale ont laissé entendre, hier, que les socialistes n'aimaient pas les entreprises. Notre position à l'égard de cet article démontre clairement le contraire. Simplement, nous défendons la justice et l'équité fiscale pour tous, à la fois pour les ménages et pour les entreprises.

L'article 3 , introduit par l'Assemblée nationale, relève d'un peu plus de 7 millions à 10 millions d'euros le seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel une PME applique le taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15

une actualisation en totalité à travers deux modifications : d'abord, en relevant la fraction de bénéfice éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 38 120 à

en deçà duquel une entreprise n'est pas assujettie à la contribution sociale sur l'IS, et en portant de 763 000 euros à 1 million d'euros le montant de l'abattement applicable.

Pour pallier cet écueil et apporter un soutien effectif à ces dernières, ma collègue Nathalie Delattre propose de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d'IS de 15 %, tout en conservant le seuil de 7,6 millions d'euros de chiffre d'affaires.

M. Jean-Marie Mizzon. En matière de solidarité plus encore que dans d'autres domaines, il faut être juste. L'effort

sur ces six amendements ? Le Gouvernement a soutenu l'introduction de cet article à l'Assemblée nationale, sur l'initiative du rapporteur Laurent Saint-Martin, avec le relèvement du seuil de 7,63 millions d'euros à 10 millions d'euros pour mieux accompagner les PME et faciliter leur développement. Il ne nous paraît pas opportun d'aller plus loin, tant sur la question du plafond de bénéfices en deçà duquel l'application du taux minoré est possible que sur celle de l'évolution du taux. Je rappelle que le Gouvernement a inscrit le taux global d'IS, c'est-à-dire non minoré,

Ainsi, les revenus de ces logements feraient l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce dispositif constitue l'une des solutions permettant de lutter efficacement contre la crise du logement, en particulier dans les zones tendues. Quel est l'avis de la commission ?

la présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement et, d'autre part, d'un remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits.

Pour ceux d'entre nous qui ne seraient pas familiers avec cette niche fiscale, je vous le dis d'emblée, elle nous coûte la bagatelle de 20 milliards d'euros,

l'avis de la commission ?

Il faut aussi que nous trouvions, ici et maintenant, les moyens de rééquilibrer les choses en France. Le dispositif proposé au travers de cet amendement vise à taxer les multinationales à hauteur de leurs bénéfices réellement réalisés en France.

l'avis du Gouvernement ?

Monsieur le ministre,

Monsieur le ministre, vous avez réussi à faire adopter une liste des territoires non coopératifs, qui est une liste nationale. Je ne vois donc pas pourquoi on ne pourrait pas retenir cette définition, d'autant que l'OCDE propose, dans son action 7, de revoir

Très concrètement, si une entreprise réalise 10 % de ses ventes en Californie, 10 % de ses profits sont taxables en Californie. Donc, cela existe !

Aujourd'hui, la déductibilité fiscale des intérêts des emprunts contractés par les entreprises est limitée à 30 % de leur résultat fiscal, conformément au dispositif prévu par la directive ATAD (), ce qui est louable dans la mesure où cette directive avait pour objectif d'empêcher un recours excessif à l'endettement. Cependant, dans le cadre de la crise que nous traversons, les résultats des entreprises sont extrêmement dégradés, et cette mesure entraîne une forte limitation de la déductibilité des intérêts et, de fait, un surcoût du financement des entreprises. Plusieurs organisations professionnelles de différents pays de l'Union européenne se sont d'ailleurs émues de cette situation auprès de la Commission et ont demandé une suspension ou une atténuation du régime pour 2020 et 2021.

Je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement sur cet amendement, qui aborde deux questions. La première est d'ordre conjoncturel : la déductibilité des charges financières est désormais plafonnée en fonction de Comment tenir compte du biais procyclique de cet encadrement, lorsque les résultats des entreprises sont dégradés, comme c'est le cas actuellement ?

monsieur le ministre, fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. En effet pour les besoins de la détermination de l'Ebitda fiscal des entreprises, la directive impose d'ajouter aux revenus soumis à l'impôt sur les sociétés, dans l'État membre du contribuable, les montants ajustés à des fins fiscales correspondant notamment à la dépréciation et à l'amortissement. et à l'amortissement. À cet égard, vous proposez de neutraliser le montant des amortissements pris en compte sur le plan fiscal, pour le calcul des plus-values ou moins-values qui majorent le résultat fiscal des entreprises concernées. Ce retraitement vise, de la même manière que pour les corrections afférentes aux reprises de provisions, à ne pas augmenter l'Ebitda au titre des deux années distinctes à raison d'une même opération. En effet, l'amortissement est ajouté au résultat fiscal pour déterminer l'Ebitda de l'année de déduction. Au titre de l'année de cession, cet amortissement est pris en compte pour le calcul de la plus-value fiscale dont il vient augmenter le montant, dans la mesure où il vient réduire la valeur d'origine du bien. Ainsi, cet amortissement tend également à augmenter le résultat fiscal pris en compte pour déterminer l'Ebitda de l'année de cession. Il convient donc selon nous, pour le calcul de l'Ebitda de l'année de cession, de retraiter le résultat fiscal en le réduisant du montant de ces mêmes amortissements, à défaut de quoi ils seraient pris en compte, à la fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été déduits et de celle au cours de laquelle l'actif a été cédé. Tel est le sens du dispositif

de nos concurrents de l'Union européenne. Et je ne parle pas de la différence, pour cette année au moins, entre les entreprises américaines et les entreprises européennes

en 2022 ! titraient voilà un an : « Le taux de marge des entreprises au plus haut depuis plus de dix ans ». Or, chaque fois que les marges augmentent, ce sont les actionnaires qui en profitent et non pas l'investissement, ou alors très peu, et surtout pas la rémunération du travail. Dans une étude datée de 2019, l'Institut des politiques publiques

Loin de relancer les investissements et les emplois, ces baisses massives n'ont fait qu'alimenter davantage la sphère financière, sous ses aspects les plus parasitaires, et l'explosion des grandes fortunes. Parallèlement, la pauvreté, elle aussi,

Cela rapporterait, ou plus exactement ne ferait pas perdre, 2,4 milliards d'euros de recettes à l'État. Au regard de tous les besoins qui seraient à financer-

est l'avis de la commission sur ces cinq amendements ? de M. Bocquet est assez classique ; il vise à réformer l'impôt sur les sociétés afin d'instaurer la progressivité de son taux en fonction du montant des bénéfices

qu'il nous paraît opportun de ne pas aller au-delà. J'ajoute à cet avis sur le fond la même remarque que celle de M. le rapporteur général sur les effets qu'aurait l'adoption de votre rédaction. Avis défavorable sur ces deux

par un dispositif d'exonération partielle d'impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation, un un minimum de quote-part pour frais et charges financières restant assujetti au taux normal de l'impôt sur les bénéfices. Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings dotées de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale fiscale très fortement décriée. De grandes entreprises ont bénéficié de cette niche. Par exemple, dès 2007, Danone a économisé 500 millions d'euros d'impôt sur les sociétés sur la cession de son pôle biscuits. En 2009, la niche a bénéficié à 6 200 entreprises, mais une dizaine d'entreprises avaient à elles seules capté 44 % du coût du dispositif. Ce coût, nous en avions connaissance à l'époque ; aujourd'hui, il est très difficile d'évaluer le coût total de la niche Copé, qui n'apparaît d'ailleurs pas clairement dans les documents d'information transmis au Parlement, ce qui pose un problème de transparence. L'estimation d'un coût annuel de 5 milliards d'euros a été avancée par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Nous vous proposons donc de supprimer purement et simplement cette niche.

légitime de prévenir la double imposition qui viendrait amputer le rendement des fonds propres investis, et réduirait l'attrait d'un certain nombre d'opérations

pour leurs bailleurs des abandons de loyers que ces derniers pourraient leur consentir dans le cadre de leur relation contractuelle. Ainsi l'État assumera-t-il une part significative de ce coût, facilitant les abandons de loyers au profit des entreprises locataires. cumulable avec les versements du fonds de solidarité, qui bénéficient directement aux entreprises locataires. Cette mesure s'inscrit dans la continuité des outils mis en oeuvre depuis le début de la crise, tels que la consécration de la déductibilité des abandons de créances locatives ou les

d'aides d'État applicable à chaque locataire, du montant du crédit d'impôt perçu par le bailleur, c'est-à-dire du seul soutien public apporté par l'État, est conforme au droit de l'Union européenne et ne fait peser aucun risque juridique sur la mesure. L'article 43 adopté en première lecture à l'Assemblée nationale met en place un régime de crédit d'impôt pour les abandons de loyers consentis, au titre de la période de confinement, au profit d'entreprises locataires qui remplissent certaines conditions. La rédaction de cet article prévoit un crédit d'impôt pour les « bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé Il est donc applicable, notamment, aux organismes privés d'HLM. Notre amendement vise, d'une part, à rattacher les dispositions de cet article à la première partie du projet de loi de finances pour 2021 et, d'autre part, à y ajouter les offices publics de l'habitat, qui ont les mêmes missions que les organismes privés d'HLM et qui louent eux aussi de nombreux locaux commerciaux, souvent situés au rez-de-chaussée d'immeubles de logements.

pour qu'il entre en vigueur dès 2020, sans attendre 2021. Trois modifications sont proposées. La première vise à étendre le périmètre des bailleurs éligibles à l'ensemble des personnes morales assujetties à un impôt sur le résultat, ce qui

aurait le mérite, comme cela a été dit, de garantir l'application immédiate du crédit d'impôt au profit des bailleurs qui acceptent d'abandonner une partie des loyers à leurs locataires.

Cet article, adopté en première partie à l'Assemblée nationale, a pour objet de déplacer les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste dans la catégorie des dépenses correspondant aux frais de production, et non plus aux frais de développement. Cette mesure ayant pour conséquence de rendre inéligibles au crédit d'impôt certaines dépenses telles que la réalisation de dossiers de presse en images ou celle de documentaires musicaux, l'article 43 du présent projet de loi a rétabli l'éligibilité de ces dépenses au crédit d'impôt et prévu l'élargissement de l'assiette du crédit d'impôt proposé à l'article 3 , qui n'a donc

Ce texte limite néanmoins le champ d'application de ce crédit d'impôt aux titres de presse présentant un caractère « d'information politique et générale ». Ce critère est très limitatif et discriminant, car il exclut la presse de la connaissance, du savoir et de l'emploi, définie, pour ce qui concerne les services de presse en ligne, à l'article 39 B du code général des impôts comme « développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique Beaucoup de ces titres comptent des abonnés à titre individuel, qu'ils soient étudiants, salariés, chercheurs ou encore retraités. Quelques exemples : les abonnés individuels

annuel destiné aux particuliers est vendu à 244 euros. Comment expliquer qu'une infirmière qui souhaite s'informer et se former sur son métier ne soit pas accompagnée dans cet effort, alors que la lectrice de l'hebdomadaire, dont

d'assujettissement à l'impôt des fonds sectoriels. Il existe des possibilités d'accompagnement, y compris à titre individuel. Toutes les mesures de bienveillance sont prises, les instructions sont données, mais nous ne souhaitons pas ouvrir de brèche dans cette doctrine. Avis défavorable sur ces deux amendements. La parole

L'article 3 est la traduction de la volonté exprimée par de nombreux parlementaires à l'occasion du PLFR 3. Le Gouvernement ne souhaite pas aller au-delà du dispositif voté à l'Assemblée nationale. J'ajoute que nous avons, en plus de ce crédit d'impôt, déployé un plan d'action pour le spectacle vivant à hauteur de 432 millions d'euros, avec des dispositions plus efficaces, car rapides, contrairement au délai qui est nécessaire pour bénéficier de l'avantage que procure un crédit d'impôt. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.

des outils pour aider le secteur culturel.

tout de suite efficients, constitueront néanmoins des leviers incitatifs très forts pour le spectacle vivant, notamment pour éviter les questions de concentration et pour aider la diversité dans son intégralité. Quel

Dans le secteur de la culture, vous le savez, il y a toutes sortes d'associations pour lesquelles ces crédits d'impôt ne seront pas totalement opérants. Or ces associations enregistrent souvent une baisse

à promouvoir l'éducation artistique de leurs enfants. pour les activités sportives. Mais dans les familles les plus modestes, qui ne veulent pas payer les cotisations alors que les cours n'ont pas lieu

au ministère, et n'aillent pas à ceux qui, dans les territoires, font vivre la culture de tous les jours

il y a aussi beaucoup d'artistes qui oeuvrent sur tous les territoires. Ce sont ceux-là, dans leur diversité, que ces dispositions viennent aider, et pas les grands établissements.

Il s'agit de copier un dispositif existant dans notre droit fiscal au bénéfice du monde agricole, celui de la dotation épargne précaution agricole. Selon les mêmes modalités, nous proposons que les propriétaires qui investissent dans la restauration de monuments classés ou inscrits puissent pratiquer la déduction fiscale qui existe déjà lorsqu'ils réalisent des travaux sur l'exercice fiscal considéré. Nous demandons qu'ils puissent bénéficier de cette déduction fiscale pour la constitution d'une provision pour travaux,

déduction qui existe déjà dans nos dispositifs de législation fiscale. Ce dispositif serait plafonné à 100 000 euros par année civile, ce qui est tout à fait raisonnable, avec quelques ajustements du plafond. En particulier, quand les monuments sont détenus par une société civile, le chiffre est multiplié par le nombre d'associés dans la limite de quatre. Par ailleurs, quand l'immeuble produit des revenus fonciers, le plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.

à développer la possibilité d'instaurer des provisions d'épargne de précaution, avec un objectif de valorisation et de restauration du patrimoine.

La déduction du revenu global proposée au travers de cet amendement ne serait subordonnée à aucune condition ni justification de difficulté avérée de la part du propriétaire du monument historique. Compte tenu du montant, cette mesure me paraît donc injustifiée. Elle est par ailleurs en contradiction avec le principe selon lequel les revenus fonciers

serait un avantage fiscal injustifié. Enfin, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) n'est pas justifiée non plus à mes yeux. Seuls les monuments historiques en sont exonérés, à la condition que les bénéficiaires de la transmission s'engagent à l'entretenir. Surtout, le placement de cette épargne de précaution me paraît pouvoir être une potentielle source d'abus puisqu'il permettrait de transmettre des liquidités en franchise d'impôt sans garantie de réalisation des travaux. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable.

Il risque même de se retrouver face à une crise de long terme due à des décalages temporels. Avec une chaîne de dépendance comme celle du cinéma, la crise actuelle des tournages va nécessairement se répercuter dans les salles sur plusieurs mois, si tant ce que chacun espère ! Cet amendement, qui vise le crédit d'impôt de production cinématographique, tend à sécuriser les tournages et,, à permettre aux salles de cinéma de bénéficier d'une programmation au moment de la réouverture. Car c'est bien sur ces deux volets, selon nous, qu'il faut agir. En effet, si les tournages sont officiellement autorisés durant le confinement, dans la réalité, les choses sont un peu plus compliquées. Premièrement, parce qu'on compte de nombreux surcoûts dus à l'achat de matériel de protection sanitaire et de tests réguliers, sans compter les limitations de personnel, entraînant des dédoublements de jours de travail ou des changements de lieu de tournage au dernier moment, par exemple. Deuxièmement, parce que les tournages peuvent aussi s'arrêter lorsqu'un cas positif se présente, ce qui s'est produit sur un tournage récemment. il faut se rappeler que ce printemps une centaine de tournages se sont arrêtés. Forcément, dans ces cas-là, les surcoûts s'additionnent pour le travail de postproduction, mais aussi les endettements liés à la préparation du film. Du côté des salles, l'enjeu est aussi double. Tout d'abord, il va falloir lever les réticences des spectateurs, ce qui impliquera une programmation riche et importante. Certes, les cinémas ont eu de la chance de pouvoir présenter le dernier film de Christopher Nolan cet été, mais qu'en sera-t-il cet hiver et au-delà ? Des reports de films attendus inquiètent la profession.

pour les oeuvres cinématographiques d'animation et les oeuvres cinématographiques autres que d'animation réalisées intégralement ou principalement en langue française, le taux est déjà de 30 %.

les toutes petites structures culturelles, suivant le spectacle, il existe une balance financière énorme entre un succès et un insuccès de participation.

Compte tenu de la crise sanitaire, investir dans les artistes en devenir sera plus coûteux : allongement prévisible de la durée des tournées, niveau d'investissements plus élevé, retours sur investissements plus longs, postes de charges en augmentation, notamment à cause des coûts sanitaires et des charges engagées pour les dates annulées ou reportées. Une bonification des taux du crédit d'impôt s'avère être un instrument simple et efficace pour le redémarrage des tournées, actuellement à l'arrêt, et l'accompagnement des entrepreneurs dans la préparation de nouvelles tournées, compromises aussi par la situation dramatique que traverse le spectacle vivant. Elle permettra, ce faisant, de protéger des centaines d'entreprises, en grande majorité de petites et moyennes entreprises, des milliers d'emplois, et de préserver la création et l'exception culturelle françaises. Cet amendement tend à remplacer le taux de 30 % par

l'avis du Gouvernement ?

particulier. Quant au mécanisme en faveur des entreprises, la loi de finances pour 2020 l'a borné jusqu'au 31 décembre 2022, et nous aurions besoin d'une évaluation complète du dispositif pour clarifier la question de l'exposition au public.

conséquent, les producteurs et les éditeurs-distributeurs dépendent des salles pour se rembourser, et ces dernières dépendent des premiers pour avoir une programmation intéressante. De plus, les producteurs dépendent des éditeurs-distributeurs pour diffuser

peuvent bénéficier, en plus de la fourniture d'un hébergement. Par conséquent, elle assimile à des investissements hôteliers les investissements affectés à une activité dont les conditions d'exercice se rapprochent des prestations fournies par un hôtel : la fourniture d'un hébergement garni de meubles et assorti des prestations habituellement proposées par des établissements hôteliers dans des conditions similaires. Cet amendement

présenté par M. Parigi,

est un dispositif qu'il convient de louer, puisqu'il a vocation à stimuler l'activité économique en exonérant les entreprises concernées de l'impôt sur le revenu ou restriction de ce mécanisme aux entreprises créées entre le 1 janvier 2019 et le 31 décembre 2020 a fortement limité le nombre d'entreprises pouvant en bénéficier, donc les retombées positives pour l'économie de l'île.

objet de permettre le cumul du dispositif avec le crédit d'impôt pour investissements, afin de créer un contexte favorable à la relance économique en Corse.

le crédit d'impôt en faveur de l'investissement en Corse existe depuis 2002. Par ailleurs, si l'on ouvrait l'éligibilité du dispositif aux entreprises installées sur le territoire avant la création des zones de développement prioritaire, cela limiterait l'aspect incitatif du zonage, du zonage, et l'aide apportée aux entreprises corses paraîtrait trop importante par rapport aux besoins d'entreprises situées dans d'autres

en Corse, pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Toutefois, sont exclus du bénéfice de ce dispositif tous les investissements déjà exploités en Corse pour des besoins de la même activité éligible.

le CIIC. Dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, la Commission européenne a assoupli les règles et la procédure relatives aux aides d'État, afin d'atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie dans l'Union européenne. En l'état, compte tenu de la situation économique post-covid, à laquelle devront faire face les entreprises insulaires, lever cette limitation pour encourager les entreprises à continuer d'investir, afin d'améliorer leur performance, serait un signal positif et encourageant pour l'économie corse.

ne peuvent concerner que des aides à finalité régionale octroyées pour un investissement initial ou pour un investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique. Il ne paraît donc pas possible d'octroyer le bénéfice du CIIC

La crise sanitaire, d'une ampleur et d'une brutalité inédites pour notre économie, impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces, immédiatement applicables : à situation

à la deuxième vague, nous vous demandons, monsieur le ministre, d'envoyer un signal positif fort aux acteurs de l'économie corse, en prolongeant jusqu'à 2025 ce dispositif et en augmentant le taux de crédit applicable à 30 % pour les PME et à 40 % pour les TPE. Nous souhaitons également que ce mécanisme puisse être étendu aux espaces commerciaux et porté à 40 % pour les entreprises ayant engagé des investissements durables et des démarches vertueuses s'inscrivant dans une logique d'économie circulaire.

En revanche, les entreprises similaires à des entreprises hôtelières qui ne sont pas des meublés de tourisme peuvent être identifiées à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, qui, eux,

Celles qui bénéficiaient déjà du crédit d'impôt bénéficieraient, avec cet amendement, d'un avantage supplémentaire,